du numérique. À plusieurs reprises depuis le mois de janvier, l’exécutif s’est dit inquiet de l’impact de la surexposition aux écrans sur la santé mentale de nos enfants. Une commission d’enquête sénatoriale et plusieurs études, dont deux rapports d’Amnesty International, ont conclu aux nombreuses conséquences néfastes de TikTok : troubles du développement cognitif, anxiété, troubles de l’attention, aggravation des tendances dépressives, depuis des années, les amendes pour non protection des données des mineurs par cette plateforme se succèdent aux États Unis, aux Pays Bas, au Royaume Uni, dans l’Union européenne. Des études scientifiques à la commission d’enquête sénatoriale, la sonnette d’alarme a été tirée à de nombreuses reprises. dernier, un comité d’experts a été missionné par le Gouvernement. Nous attendons leurs conclusions de manière imminente. Pourtant, nous savons qu’il existe déjà des solutions. Certaines ont d’ailleurs été évoquées jusqu’au sein de l’exécutif, notamment la régulation de l’usage des écrans et l’interdiction effective effective de TikTok. Madame la secrétaire d’État, il est urgent d’agir. Pouvez vous nous présenter l’état des réflexions et les premières pistes envisagées par le comité d’experts ? Allez vous vous battre pour imposer ce sujet à l’échelon européen, puisque la France ne peut pas interdire ou bloquer seule des plateformes ? De quels outils notre pays dispose t il pour faire respecter des mesures de blocage ou de limitation d’accès ? Enfin, qu’allez vous faire pour former les adultes, qui, souvent, n’ont pas les moyens d’apprendre aux enfants un bon usage du numérique ? La parole

Tout d’abord, à l’échelon européen, la France a été un fer de lance dans l’adoption du règlement européen sur les services numériques, dit (DSA). À ce titre, TikTok a désormais – vous le savez – l’obligation d’analyser et de prendre les mesures nécessaires face au risque systémique susceptible d’avoir des conséquences négatives graves sur le bien être physique et mental des mineurs. Le DSA prévoit également l’audit des algorithmes qui gouvernent ces plateformes par des régulateurs ou des tiers

des applications sur smartphone. Le Président de la République a par ailleurs lancé une commission « écrans » composée d’experts. Elle est chargée de remettre des propositions structurantes d’ici à la fin de ce mois ; nous les attendons. À ce stade, je n’ai pas encore les conclusions et je ne peux donc pas vous livrer les pistes qui sont explorées. Toutefois, vous pouvez compter sur mon engagement plein et sur celui du Gouvernement pour une régulation responsable de nos réseaux sociaux et pour maintenir des discussions exigeantes avec ces acteurs également – vous avez raison – à l’échelon européen. La parole est à Mme Agnès

En effet, dans le département du Doubs, et dans le cadre de l’élaboration du volet routier du contrat de plan État région 2023 2027, le conseil départemental envisage de répondre favorablement à la sollicitation de l’État pour accepter une délégation de maîtrise d’ouvrage portant sur l’aménagement de la route nationale 57 (RN57) à l’entrée sud de Pontarlier. délégation de maîtrise d’ouvrage a été réaffirmée par l’article 41 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de loi 3DS, permettant par là même de faciliter l’inscription de ces opérations dans les contrats des plans État région en limitant le montant au montant hors taxe des investissements au motif de l’éligibilité des dépenses départementales correspondantes au FCTVA.

1615 13 du code général des collectivités territoriales, les collectivités ne peuvent désormais plus bénéficier du FCTVA pour les investissements qu’elles réalisent dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage sur le domaine public routier de l’État.

l’article 41 de la loi 3DS, l’État peut confier à un département la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant un caractère prioritaire. Ce montage juridique, sans s’y assimiler, s’apparente à une délégation de maîtrise d’ouvrage et les dépenses exposées doivent être enregistrées à des comptes d’opération pour compte de tiers, plus précisément au compte 4581. Dans le cadre de la réforme de l’automatisation du FCTVA, les travaux réalisés pour le compte de tiers ne sont plus éligibles à ce dernier. Dans le cas particulier des opérations réalisées dans le cadre des délégations de maîtrise d’ouvrage visées par la loi 3DS, les dépenses sont remboursées par l’État dans les conditions prévues par voie de convention. Pour autant, cela n’exclut pas la possibilité, pour la collectivité mandataire, de contribuer au financement de l’opération, en particulier si elle souhaite réaliser des travaux supplémentaires. Sa contribution s’apparente à un fonds de concours et est traitée comme une subvention d’équilibre de l’opération sous mandat. Or le département bénéficiera du FCTVA au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement qu’il effectue sur le domaine public routier national.

d’équipement à l’État – Voirie » et au crédit du compte 4582 par opération d’ordre budgétaire. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que ces écritures d’ordre budgétaire ne font pas encore l’objet d’un traitement automatisé. Aussi, la collectivité doit procéder à la déclaration de cette dépense par l’intermédiaire d’un état manuel pour bénéficier du FCTVA.

ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue en Île de France. Le produit de cette taxe a vocation à être reversé à Île de France Mobilités, dont les besoins de financement à court et à moyen termes sont très importants. Cette nouvelle taxe additionnelle s’ajoute – il faut le rappeler – à celle qui avait été prévue par la loi de finances pour 2019, au taux de 15 %, et qui bénéficie à la Société du Grand Paris, devenue Société des grands projets en 2023. Le moins que l’on puisse dire, c'est que le législateur a eu la main particulièrement lourde. Le mécontentement des élus locaux essonniens est grandissant, car ces deux instruments fiscaux ont des répercussions directes sur la fréquentation de leurs hébergements touristiques. publics de coopération intercommunale (EPCI) de l’Essonne situés aux confins de l’Île de France, qui se trouvent confrontés à la concurrence directe des régions voisines, où cette nouvelle taxe additionnelle ne s’applique pas. Comble de l’absurdité, les établissements hôteliers et les chambres d’hôtes concernés pratiqueront une taxe de séjour plus élevée qu’à Nice, Saint Tropez ou Avoriaz ! Il est bien entendu impensable que les collectivités territoriales suppriment la taxe de séjour à laquelle la taxe additionnelle est adossée, car elles mènent des politiques actives en faveur du tourisme vert ou de la protection de leurs espaces naturels. Une adaptation législative est, par conséquent, nécessaire. Elle est d’autant plus urgente que ces territoires de l’Essonne éloignés de la métropole parisienne ne bénéficient pas, ou très peu, des services offerts

vous faites état d’une situation, celle de la couverture du département de l’Essonne par le réseau de transport francilien, à laquelle l’instauration de la taxe additionnelle à la taxe de séjour, pour le financement d’Île de France Mobilités, a justement vocation à remédier. À l’image de la récente mise en service de la ligne tram train T12, T12, l’offre de transport en Île de France va profondément évoluer. Il en résulte un besoin accru de financement pour Île de France Mobilités afin de soutenir les réalisations déjà entreprises et renouveler impérativement le matériel roulant. L’instauration de cette taxe additionnelle à la taxe de séjour fait suite à la signature, le 26 septembre dernier, entre l’État et Île de France Mobilités, d’un protocole pour financer les transports en commun franciliens. Cet accord doit garantir une stabilité des moyens sur la période.

Cette taxe additionnelle, dont le taux a fait l’objet d’une concertation avec les représentants de l’hôtellerie, doit rapporter 200 millions d’euros par an. Cela permettra d’aligner la région capitale sur les standards de contribution du tourisme d’autres capitales européennes. Enfin, la distorsion de concurrence que vous redoutez, entre les hébergements situés en Essonne et ceux qui sont situés en région Centre Val de Loire, semble très limitée eu égard au montant de la surtaxe par nuitée, en particulier pour la clientèle d’affaires présente dans le département de l’Essonne. Toutefois, un bilan sur le rendement et les effets de la surtaxe pourra être dressé après une année d’application pour que nous puissions éventuellement corriger les choses. La

La consécration du choix durable du recours à cette énergie semble désormais actée dans l’article 1 de l’avant projet de loi sur la souveraineté énergétique. Pour parvenir à une production d’électricité supplémentaire, il est prévu de faire construire six EPR2 par EDF pour une mise en service théorique d’ici à 2035, ainsi que de lancer des études pour la création de huit autres EPR2, produisant au moins 13 gigawatts. D’ores et déjà, trois sites ont été retenus pour la première tranche de nouveaux réacteurs : Penly, Le Bugey et Gravelines. Il reste donc à déterminer les sites accueillant les installations de la deuxième tranche. Dans ce cadre, le CNPE de Golfech, seul site nucléaire en Occitanie, possède, je le crois, de solides atouts en termes de sûreté, d’infrastructures nécessaires, de potentiel de production d’électricité, de compétences techniques et humaines pour accueillir deux réacteurs de nouvelle génération. Dès lors, je souhaite connaître les intentions du Gouvernement

Mme la secrétaire d’État. Monsieur le sénateur Bonhomme, vous l’avez rappelé, la stratégie énergétique du Gouvernement, dont le Président de la République a donné le cap à Belfort en février 2022, repose sur quatre piliers pour permettre à la France de sortir des énergies fossiles : la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique, le déploiement des énergies renouvelables

de Penly, de Gravelines et du Bugey. Nous étudions actuellement la construction de huit réacteurs additionnels. Nous souhaitons pouvoir en tirer les conclusions dans les toutes prochaines années. En tout état de cause, l’année 2023 a permis d’adopter la loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants.

un fournisseur d’électricité et celui auquel l’électricité est revendue. Nous avons constaté ces derniers mois une forte hausse des prix sur le marché de l’électricité, nécessitant même une intervention de l’État pour soulager les consommateurs. Dans un secteur ouvert à la concurrence, le prix de revente dépend de la valeur du marché. Pourtant, les particuliers producteurs d’électricité, notamment ceux qui sont équipés de panneaux photovoltaïques, se voient racheter leur surplus électrique à un prix dérisoire. Ils sont contraints d’accepter une valorisation en dessous du prix de revente aux consommateurs, en raison de la position dominante des fournisseurs d’énergie, EDF dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui. Il est inacceptable que certains particuliers revendent le kilowattheure à 10 centimes d’euros quand celui ci

les particuliers qui installent des panneaux photovoltaïques ont, le plus souvent, recours à l’autoconsommation. Et lorsqu’ils produisent à certains moments plus qu’ils ne consomment, ils peuvent – vous l’avez dit – réinjecter dans le réseau le surplus d’électricité. Cette quantité d’électricité est payée à un tarif fixé par arrêté, établi pour couvrir une rémunération normale de l’investissement réalisé. Le Gouvernement ne souhaite pas encourager les comportements spéculatifs sur la volatilité des prix de gros, autant pour les fournisseurs d’énergie que pour les particuliers. Comme vous le savez, la hausse des prix de l’énergie que l’Europe a connue en 2022 et 2023 est le résultat malheureux de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Elle a nécessité le déploiement de moyens budgétaires colossaux pour protéger nos consommateurs. Dans ces circonstances, l’autoconsommation s’est révélée particulièrement protectrice en complément. C’est pourquoi le Gouvernement a tenu à maintenir les différents dispositifs de soutien,

sont utilisées pour de l’autoconsommation, soit une multiplication par six de l’énergie photovoltaïque autoconsommée depuis quatre ans, avec une croissance de 84 % entre 2022 et 2023. Dans sa stratégie énergétique, le Gouvernement s’appuie sur un déploiement important de l’autoconsommation,

plus vertueuses pour la préservation de la ressource en eau par le développement et l’accompagnement des filières agricoles viables, afin d’adapter le territoire au changement climatique. Il s’agit, par exemple, de l’agroforesterie, du maintien des prairies ou de leur remise en état, du développement de l’agriculture biologique. Les agriculteurs vont ainsi modifier leurs pratiques afin de réduire la pression de pollution par les produits phytosanitaires sur les aires d’alimentation de captage d’eau potable classées prioritaires pour la métropole du Grand Paris.

À cet égard, la politique agricole commune (PAC) constitue un des leviers principaux. Le plan stratégique national, approuvé par la Commission européenne, montre un soutien important aux exploitants agricoles dans leur transition agroécologique, avec notamment la création de l’écorégime. Il s’agit d’une aide versée aux exploitants agricoles qui s’engagent volontairement à mettre en place, sur l’ensemble de leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement. L’objectif de l’écorégime, versé à l’hectare et par exploitation, est d’accompagner est d’accompagner les agriculteurs dans leur transition en massifiant ces pratiques. Cette massification est permise par l’identification de trois voies d’accès distinctes : celle des « pratiques », celle de la « certification environnementale » et celle des « éléments favorables à la biodiversité L’écorégime est assimilable à un dispositif du type paiements pour services environnementaux, avec des moyens financiers importants. En effet, l’écorégime représente 25 % des aides directes du premier pilier de la PAC, soit plus de 1,7 milliard d’euros par an.

ne sont pas cumulables avec les Maec, c’est parce qu’ils sont susceptibles de financer les mêmes pratiques. Dans le cadre d’un PSE, comme dans celui des Maec, un exploitant s’engage à respecter un certain nombre d’obligations, qui peuvent se recouper. L’enjeu est donc d’articuler ces dispositifs de PSE et les aides de la PAC, afin qu’il n’y ait pas de double financement.

Si je comprends bien, sur ce programme innovant et singulier, qui mobilise un territoire rural et la métropole du Grand Paris, il ne pourra pas y avoir de cumul

Comme l’an dernier à la même époque, cette académie – c’est plus particulièrement le cas dans le département de la Haute Vienne – subit une véritable saignée dans le premier degré : dix huit suppressions de postes, vingt neuf fermetures de classes et aucune création de poste dans la brigade de remplacement déjà exsangue. On va sûrement m’opposer la baisse des effectifs et la baisse démographique… Mais les chiffres ne peuvent pas tout expliquer ! Dans mon département, par exemple, le nombre de professeurs par élèves est inférieur à la moyenne nationale et à la moyenne académique. Ce chiffre là, les services du ministère En Haute Vienne, comme dans de nombreux autres départements, la carte scolaire est vécue chaque année comme un couperet. Sur le fond comme sur la forme, elle suscite toujours plus de critiques. Si l’éduction nationale est vraiment une priorité, il faut donner aux enseignants les moyens d’exercer leur métier dans de bonnes conditions. À l’heure où le Gouvernement annonce de nouvelles restrictions budgétaires, nous ne pouvons pas accepter de sacrifier l’avenir de nos enfants sur l’autel de la rigueur ! Purement arithmétique, sans prospective, ni perspective d’ailleurs, la carte scolaire telle qu’elle est élaborée aujourd’hui est inadaptée. Pourquoi ne pas revoir la méthode en introduisant, par exemple, une vision pluriannuelle ? Mme Belloubet l’a d’ailleurs évoqué le 14 février dernier, lors de la séance des questions d’actualité au Gouvernement. Pourquoi ne pas mieux associer les maires, les élus ? L’an dernier déjà je plaidais ici même pour un moratoire, afin de nous donner le temps de la réflexion. Il n’est pas trop tard. Le Gouvernement doit entendre la colère et les inquiétudes dans nos territoires et remettre l’école publique, laïque et républicaine au centre de nos villages comme de nos villes !

Des réponses adaptées aux territoires ruraux ont été élaborées au cours des dernières années. Je pense à l’allocation progressive des moyens, qui tient compte de l’indice d’éloignement, ou encore au dispositif des territoires éducatifs ruraux.

le budget 2024 de l’éducation nationale et de la jeunesse est, et demeure, le premier budget de la Nation. Dans le premier degré, compte tenu de la baisse démographique déjà évoquée à la rentrée 2024, la réduction du nombre d’emplois dans le public n’empêchera en rien la poursuite

en 2017, en accueillera 21,5 en 2023. Ce chiffre devrait encore diminuer pour atteindre son plus bas niveau historique à la rentrée 2024. Le Gouvernement sera donc au rendez vous des priorités pour l’école primaire achèvement du dédoublement des grandes sections de maternelle en éducation prioritaire, progression de la scolarisation en très petite section des enfants de 2 ans dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,

C’est le cas à Philippsbourg, mais aussi au sein des écoles du regroupement pédagogique intercommunal dispersé (RPID) de Voyer, Hermelange et Nitting, ou encore dans la commune de Wittring. Sans surprise, cette situation est incompréhensible pour les élus mosellans de ces communes rurales, qui trouvent hautement contestables les estimations aboutissant à ces résultats. Les enfants mosellans sont des citoyens à part entière. Ils n’ont pas à pâtir d’un éloignement géographique des grands centres urbains. Comment ne pas s’étonner de décisions en totale contradiction avec les annonces gouvernementales

À la rentrée 2023, 18 % des élèves étaient scolarisés dans l’une des 14 802 écoles publiques situées en zone rurale. Toutefois, il ne peut y avoir de réponse unique à la diversité des situations : si certaines de ces écoles connaissent des difficultés d’accessibilité, d’autres bénéficient de la réussite des projets de regroupement pédagogique qui sont conduits. Les taux d’encadrement y sont globalement favorables, avec 19,9 élèves par classe dans les communes rurales éloignées et 21,6 dans les communes rurales périphériques, soit une moyenne inférieure au ratio national, hors éducation prioritaire. La réforme de l’allocation des moyens d’enseignement du premier degré public, mise en œuvre depuis la rentrée 2015, a permis de prendre en compte la difficulté sociale et le contexte territorial. Cette évolution favorable a été confortée par l’engagement pris, depuis la rentrée scolaire 2019, de ne fermer aucune école rurale sans l’accord du maire. dans un contexte de baisse démographique – 5 340 élèves en moins dans les écoles publiques du premier degré entre les rentrées 2017 et 2023 –, le taux d’encadrement est passé de 5,45 à 5,86. Il devrait de nouveau augmenter à la prochaine rentrée

Dans les communes rurales de Moselle, ce taux d’encadrement tombe à 20, très proche de la moyenne nationale. Dans les communes rurales, il est de 21,4, soit plus favorable que la moyenne nationale, tandis que dans les zones urbaines denses, il s’élève à 22,1. Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour que tous les élèves, quel que soit leur territoire,

souffrent d’exceptions. Il y a, dans ces écoles, un taux d’encadrement insuffisant. C’est la raison pour laquelle je vous demande instamment de reconsidérer l’approche

Contestable sur la forme, ce licenciement l’est encore plus sur le fond : il semble dû à la participation de cet employé à une grève contre la réforme des retraites. Plusieurs autres facteurs précaires sont dans la même situation, qui s’apparente à un non respect flagrant du droit de grève. Ce licenciement en dit long sur l’évolution du métier de facteur, de plus en plus ubérisé. Ainsi, pour les nouvelles embauches, La Poste n’offre plus le statut de facteur, mais recourt à des intérimaires, des sous traitants ou des CDI en contrats « groupements d’employeurs logistiques » (GEL). Ces contrats

À travail égal, les salariés en contrat GEL ont des paies plus faibles, ne touchent pas les primes, n’ont pas droit aux formations ou au maintien de salaire pour s’occuper ponctuellement de leurs enfants. La Poste a donc un système à deux vitesses, qui lui permet de faire des économies et de diviser les salariés pour empêcher qu’ils ne se coordonnent. C’est justement pour éviter ce scénario qu’il est normalement interdit de recourir à ces contrats pour « un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise », une règle violée par La Poste.

Face à ces pratiques visiblement illégales, le syndicat Sud PTT prépare une plainte pour prêt illicite de main d’œuvre et marchandage, et a alerté l’inspection du travail. En attendant des suites judiciaires, comment accepter que La Poste, propriété de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations, qui reçoit 500 millions d’euros de subvention par an et réalise des bénéfices, s’adonne à de telles pratiques ?

il ne m’appartient pas de commenter des procédures judiciaires en cours. Toutefois, je peux vous rappeler l’état du droit. Vous avez évoqué le licenciement d’un travailleur temporaire mis à la disposition du groupe. Sans statuer sur l’éventuel caractère abusif de cette décision, je vous indique qu’une entreprise de travail temporaire doit proposer au salarié, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours. À défaut, elle doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat.

peut bien sûr saisir les prud’hommes. Vous contestez le recours par La Poste à des salariés d’un groupement d’employeurs et alléguez une méconnaissance du principe d’égalité de traitement. Ce groupement ne respecterait pas non plus le principe de non lucrativité de son activité. La loi autorise les groupements d’employeurs, afin de mettre des salariés à disposition de leurs membres. Les contrats de travail conclus par le groupement doivent garantir l’égalité de traitement en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale

le déficit important de France Compétences a justifié des baisses drastiques de la prise en charge du coût de formation qui touchent d’abord les métiers de l’artisanat, pour lesquels ces coûts sont incompressibles.

Madame la ministre, quels sont les moyens prévus par le Gouvernement pour garantir la soutenabilité des coûts de formation des apprentis dans les métiers dont la France a besoin ?

l’apprentissage constitue une réponse efficace aux tensions de recrutement que nous connaissons partout sur le territoire, y compris dans l’artisanat, historiquement tourné vers cette voie d’entrée dans les métiers.

Par ailleurs, grâce à son opérateur France Compétences, l’État est chargé d’assurer un travail de régulation des niveaux de financement de l’apprentissage. Ce travail repose sur l’analyse

de garantir un juste niveau de financement au regard des coûts réels constatés. Lorsque les niveaux de prise en charge des coûts contrats ont été revus en 2022 et 2023, les règles des procédures pour les déterminer ont été les mêmes

Pourtant, dans le Val d’Oise, l’un des territoires les plus jeunes de France métropolitaine, les moyens manquent. Le secteur comprenant la ville de Cergy Pontoise et une partie du Vexin rencontre d’immenses difficultés. Seuls deux médecins répondent aux besoins d’une population de 68 000 mineurs dans onze unités d’amont et d’aval. À Argenteuil, ville de 110 000 habitants, les actions déployées en pédopsychiatrie sont assurées par 1,6 équivalent temps plein. Ces effectifs sont largement insuffisants, dans un territoire où les demandes de consultations et de prises en charge ne cessent d’augmenter, en particulier depuis la pandémie de covid Les délais de demande de rendez vous deviennent infernaux pour les familles. Les places dans les établissements médico sociaux sont bien trop rares. Dans ce secteur, 600 enfants attendent pour entrer en institut médico éducatif (IME). Comment les accompagner au mieux et leur permettre de s’épanouir ?

qui assurait un suivi médico psychologique de jeunes souffrant de troubles psychologiques et psychotiques. La psychiatrie et la pédopsychiatre sont les parents pauvres de notre système de santé. Madame la ministre, quels moyens humains et financiers seront mis en œuvre pour assurer la continuité de ce service public et répondre à votre priorité gouvernementale dans le Val d’Oise ? Bravo

en place pour attirer les professionnels de santé dans le département. Je pense à l’amélioration de leurs conditions de travail, à l’attribution d’aides ciblées pour les internes ou encore au cofinancement des initiatives des établissements publics en faveur du logement de leur personnel soignant. Par ailleurs, l’amélioration de la prise en charge des Franciliens en santé mentale, en particulier des plus jeunes, constitue une priorité d’intervention du nouveau projet régional de santé de l’ARS d’Île de France. En 2023, le département du Val d’Oise, reconnu prioritaire, a ainsi pu bénéficier de 800 000 euros de financement pour les trois projets majeurs venant renforcer l’offre en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Enfin, concernant l’accompagnement des enfants en situation de handicap, pour lesquels vous connaissez mon engagement, l’ARS a lancé le 12 octobre 2023 le plan Inclus’IF 2030, financé à hauteur de 310 millions d’euros par la région.

Ma région, en particulier mon département du Nord, compte peu de fleuves et de rivières ; l’eau est puisée essentiellement dans les nappes phréatiques. L’eau du robinet est l’un des éléments les plus surveillés et contrôlés.

Certains d’entre eux, comme le nitrate et autres pesticides, sont très connus, mais de nouveaux polluants, appelés métabolites, font désormais l’objet d’une attention particulière des autorités sanitaires.

l’un de mes déplacements dans le Nord, dans l’arrondissement de Douai, j’ai rencontré des gestionnaires d’eau potable. Ils sont contraints de réaliser de savants mélanges de captage d’eau pour essayer d’obtenir des résultats satisfaisants, qui peuvent malgré tout dépasser les taux autorisés tout en étant déclarés conformes à la consommation. Cette situation conduira les gestionnaires d’eau potable à investir dans des usines de traitement onéreuses, afin de poursuivre l’exploitation des ressources dont ils ont la charge. Madame la ministre, compte tenu de cette situation, je souhaite connaître la politique que le Gouvernement compte mettre en place afin d’accompagner les gestionnaires d’eau potable.

Pour les métabolites de pesticides, des consignes nationales ont été établies en 2010, puis mises à jour en 2020, 2022 et 2023. La réglementation européenne fixe une limite non sanitaire, mais de qualité, à 0,1 microgramme par litre. En cas de dépassement et en tenant compte d’un principe de proportionnalité, les États peuvent fixer une valeur sanitaire en deçà de laquelle, par dérogation, la consommation d’eau demeure possible. Un plan d’actions interministériel a été acté en octobre 2023. Tout en maintenant la distribution de l’eau, il vise notamment à informer de manière transparente la population, à accélérer l’expertise sanitaire des agences pour définir des valeurs de référence lorsque celles ci n’existent pas,

est bien sûr d’étendre la surveillance à d’autres pesticides. À ce titre, le Gouvernement a demandé au Haut Conseil de la santé publique de proposer des mesures proportionnées de gestion des risques

employant moins de 350 agents, des missions de gestion, d’assistance et d’expertise dans le domaine des ressources humaines. Ils sont donc très précieux pour les élus locaux. Les centres de gestion coopèrent également entre eux à l’échelon régional, en mutualisant plusieurs de leurs missions dans un souci d’efficacité et d’économie de leurs moyens. En Normandie, cette coopération est particulièrement efficace et bien adaptée aux problématiques relatives aux ressources humaines que partagent les maires et les présidents d’intercommunalité. Les CDG se sont par ailleurs volontairement regroupés à l’échelon national au sein d’une association, la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), qui assure leur représentation auprès du Parlement, du Gouvernement ou des administrations centrales et coordonne certaines de leurs missions. Au cours des dernières années, plusieurs tentatives de fusion régionale ou nationale des centres de gestion ont été entreprises par les pouvoirs publics, à contre courant, il faut le souligner, des besoins de proximité exprimés par les élus employeurs. Aujourd’hui, dans le Calvados comme ailleurs, une majorité de CDG se mobilisent de nouveau pour repousser la transformation de leur fédération en établissement public national, ce projet faisant poindre le risque d’une mise sous tutelle, puis, à terme, de leur disparition au profit d’une structure nationale déconcentrée, pilotée depuis Paris. Les élus des centres de gestion considèrent que le statut associatif actuel de la FNCDG donne satisfaction. Aussi, je souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière et savoir s’il compte prendre en considération les positions exprimées

indispensable de ces établissements publics, qui assurent, pour le compte des collectivités territoriales et leurs établissements, des missions essentielles en matière de gestion des ressources humaines. Je le dis d’autant plus volontiers que j’ai moi même siégé au sein de Vous faites état de l’inquiétude de certains centres de gestion quant à une possible transformation de la Fédération nationale des centres de gestion en établissement public national. Le Gouvernement tient à rappeler la place essentielle de la FNCDG, partenaire et interlocuteur partenaire et interlocuteur de longue date sur tous les sujets de recrutement et de gestion des personnels territoriaux. Son rôle de représentation, d’animation et de coordination des centres de gestion est primordial. de gestion est primordial. La FNCDG a certes conduit une réflexion sur le sujet de sa transformation en établissement public national, réflexion qui a connu sa conclusion lors de son assemblée générale du 7 décembre dernier, durant laquelle il a été décidé de ne pas poursuivre ce projet.

telle transformation, qui relèverait en outre du domaine de la loi, n’est pas non plus à l’ordre du jour du Gouvernement. J’espère que cette réponse vous aura rassurée, madame la sénatrice. La parole

une organisation qui donne toute satisfaction sur nos territoires ? Les élus de mon département qui m’ont interpellée à ce sujet seront, je pense, satisfaits de votre réponse.

Frontalier de la Suisse, plus particulièrement de la métropole genevoise, ce territoire est confronté à une problématique majeure de cherté de la vie. À titre de comparaison, les prix du logement y sont pratiquement au même niveau qu’en Île de France. Cela a de graves conséquences pour pour les fonctionnaires, certains se retrouvant dans des situations de grande précarité, et pour les collectivités, qui peinent à recruter afin d’assurer le bon fonctionnement de leurs services publics. Depuis 2020, j’ai interpellé à plusieurs reprises le Gouvernement sur ce sujet

de Haute Savoie et du Pays de Gex, à la suite de la mobilisation de nombreux parlementaires locaux. Même si le montant de cette indemnité reste modique, environ 50 euros net par mois en moyenne, c’est une première avancée.

alors même que les problématiques de vie chère sont les mêmes dans tout le territoire. C’est incompréhensible pour nos élus ! Ce périmètre restreint entraîne une rupture d’équité : d’une part, du côté des agents, qui ne bénéficient pas tous de cette indemnité, bien qu’ils soient tous confrontés aux coûts exorbitants des logements ; d’autre part, du côté des collectivités, celles qui ne bénéficient pas de l’indemnité de résidence subissant un déficit

Pour rappel, celui ci vise à attribuer un complément de rémunération à certains agents selon la commune où ils exercent leurs fonctions pour compenser les disparités du coût de la vie. Vous le savez, cette indemnité est fondée sur un zonage qui date de 1962, en décalage avec la situation économique actuelle. Cependant, sa mise à jour serait très complexe. Pour autant, nous devons apporter des réponses, tant pour compenser les coûts liés au logement que, de manière plus générale, pour favoriser l’attractivité de certains territoires. Ce dernier enjeu est au cœur de l’agenda social mis en place par le ministre de la transformation et de la fonction publiques et du projet de loi sur la fonction publique

particulière sur le marché immobilier et sur le marché de l’emploi public local : c’est ce qui nous a conduits à créer au mois de décembre 2023 une indemnité de résidence spécifique au taux maximum de 3 %, une mesure qui était attendue depuis longtemps.

de créer de nouveaux leviers d’intervention. Avec le comité interministériel pour le logement des agents publics (Cilap) et la délégation interministérielle dédiée, nous améliorons l’accès des fonctionnaires aux dispositifs d’aide au logement

sceaux, ministre de la justice. Madame la ministre, j’alerte de nouveau le Gouvernement sur le projet de construction d’une prison à Noiseau, dans le Val de Marne. L’orientation du Gouvernement est connue : il a engagé cinq nouveaux projets pénitentiaires en Île de France, mais l’essentiel des nouvelles places est concentré sur le site envisagé à Noiseau – 30 % des places se trouveront dans ce village de 4 700 âmes. Le 1 février dernier, M. Patrick Farcy, maire de Villecresnes et conseiller départemental du Plateau briard, a adressé un courrier à M. le Premier ministre dans lequel il rappelait de façon limpide l’ensemble des problèmes soulevés par ce projet, je le rappelle, l’opposition de l’ensemble des élus locaux, toutes tendances politiques confondues. D’abord, ce projet s’insère dans un département qui est déjà fortement marqué par un site pénitentiaire, celui de Fresnes, deuxième plus grand centre pénitentiaire de France, dont les besoins de mise en conformité sont criants et pour lesquels l’État a déjà été condamné. Ensuite, la construction éventuelle de cette prison reviendrait à remettre en cause 50 hectares de terres agricoles fertiles encore exploitées. Avec elles, je vous parle de la destruction d’une zone humide essentielle, abritant une nappe phréatique fragile, ainsi qu’une biodiversité riche accueillant des espaces rares.

cinq sites potentiels qui ont été examinés pour ce projet en Île de France, les études foncières menées depuis des années ont bien entendu porté d’abord sur des friches industrielles.

posant des problèmes de sécurité. Certes, le projet engendrera une diminution de foncier agricole, mais il sera conçu pour limiter au maximum ses impacts sur le milieu agricole. L’Agence publique pour l’immobilier de la justice (Apij), qui assure la maîtrise d’ouvrage du projet, prendra contact avec les deux exploitants agricoles concernés afin d’évaluer précisément l’impact sur le fonctionnement de leur exploitation et d’adapter si besoin le projet pour le limiter. À ce jour, les ce jour, les informations obtenues sur l’exploitation de M. Naudier sont les suivantes : sur 199 hectares, seuls 13 seraient utilisés par l’établissement pénitentiaire. Une étude préalable sera lancée prochainement afin de définir les mesures compensatoires. L’existence d’un ancien réseau de drainage sous terrain sur le site d’implantation du projet est connue. L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a été désigné et les dates de son intervention seront définies prochainement. Concernant les risques d’inondation, une entreprise spécialisée a d’ores et déjà été sollicitée pour réaliser un état des lieux. J’en viens au trafic routier. Le Gouvernement a pris note des fortes inquiétudes, notamment sur les conditions de circulation très dégradées de la route départementale 136. Une étude de mobilité et des flux sera diligentée. Elle prendra en compte le projet d’agroquartier développé par les collectivités avoisinantes. Sans attendre ces résultats, il a d’ores et déjà été retenu la création d’un accès secondaire à l’établissement le chemin de la croix Saint Nicolas, dédié aux véhicules légers, afin d’éviter une concentration des flux sur la RD 136, déjà

et des outre mer. Madame la ministre, l’humusation est un mode de sépulture qui se veut plus respectueux de l’environnement que les deux modes actuellement autorisés en France : l’inhumation et la crémation. Ce processus vise à réintégrer le corps humain dans le cycle du vivant en transformant le corps du défunt en humus, qui est la couche supérieure du sol créée par la décomposition de la matière organique. La légalisation de l’humusation fait l’objet de revendications dans notre pays. est effective dans six États des États Unis d’Amérique, mais dans aucun pays européen. En 2016, le ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve avait évoqué la nécessité de mener une réflexion approfondie sur le sujet, en collaboration avec le Conseil national des opérations funéraires

Elle pourrait être en outre une solution économique, car elle n’engendre pas de frais de concession. Madame la ministre, le Gouvernement compte t il mener une réflexion sur la question, notamment en étudiant sa faisabilité d’un point de vue sanitaire,

L’humusation, qui consiste à transformer les corps en humus, soulève un certain nombre de questions légitimes et nécessite une réflexion et une concertation approfondies, notamment dans ses aspects éthiques, sociétaux et environnementaux. Le statut juridique des particules issues de l’humusation, et sa compatibilité avec l’article 16 1 1 du code civil – « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » –, doivent notamment être étudiés. Vous souhaitez savoir si le groupe de travail prévu par le Gouvernement a été enterré… plaisir de vous dire que tel n’est pas le cas. Il sera constitué avant la fin du premier semestre 2024, sous l’égide du Conseil d’État, afin d’examiner les possibilités d’évolution de la réglementation sur ce sujet. Il réunira des parlementaires, des universitaires, des représentants des collectivités territoriales, des opérateurs funéraires et des familles, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des administrations concernées. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour la réplique.

C’est faire face immédiatement, dès son arrivée, aux carences d’un État qui a oublié sa mission consistant à garantir l’accès aux droits fondamentaux prévus par la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Les personnes primo arrivantes sont confrontées à une absence d’organisation pour le premier accueil et à la baisse des moyens que vous y consacrez. Le nombre de personnes prises en charge par l’État dans le cadre des mises à l’abri dédiées aux migrants en rue est passé de 12 154 en 2017 à 4 105 en 2023 à Paris. Si, en 2015, cette désorganisation pouvait s’expliquer par la hausse rapide des arrivées, depuis neuf ans, la politique mise en place par votre gouvernement n’a jamais permis un premier accueil et une prise en charge digne des personnes arrivées. Elle n’a jamais eu comme ambition de faire disparaître les grands campements, souvent situés dans le Nord Est parisien. Deux périodes font exception : lorsque la bulle humanitaire, créée à la demande de la maire de Paris, Anne Hidalgo, a fonctionné et lors de la crise sanitaire et des confinements. C’est la preuve que lorsque la volonté est là, cela fonctionne et que rien n’est inéluctable. Depuis la fin de la crise covid, des centaines de personnes primo arrivantes vivent de nouveau dans une extrême précarité. Hier, plus de 400 jeunes, évalués majeurs par le département de Paris et non pris en charge depuis des mois par l’État, ont été expulsés par la préfecture de police, sans aucune solution d’hébergement, même transitoire, malgré les demandes des élus parisiens. Face aux lacunes de l’État, la Ville de Paris se mobilise et héberge ces familles, ces femmes, ces hommes 436 personnes dans des gymnases municipaux, début février. Plus récemment, la municipalité a dû ouvrir un lycée pour héberger des familles, dont les enfants scolarisés dans nos écoles, dormaient, pour beaucoup, également dans des écoles, grâce à la solidarité sans faille des communautés éducatives.

Je me permettrai d’opposer d’autres chiffres à ceux que vous avez cités. La situation des personnes primo arrivantes en situation de rue est suivie de près par la préfecture de la région Île de France, qui mène régulièrement, en lien avec la préfecture de police de Paris, des opérations de mise à l’abri. En 2023, 35 opérations ont ainsi pu être conduites, contre 19 en 2022. Ces opérations, qui concernent les personnes en situation de rue, quelle que soit leur situation administrative, ont permis de mettre à l’abri 6 500 personnes. Pour contrebalancer le regroupement des demandeurs d’asile en Île de France, le Gouvernement met en œuvre depuis 2021 une politique d’orientation de ces personnes vers des lieux de prise en charge dans les différentes régions. régions. Plus de 61 000 personnes se sont ainsi vu proposer une orientation vers un hébergement en région par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) depuis la mise en place du dispositif. En outre, le Gouvernement a mis en place au mois d’avril 2023 dix sas d’accueil régionaux destinés à accueillir les personnes sans solution d’hébergement à l’issue d’opérations de mise à l’abri, le temps d’examiner leur situation sociale et administrative avant de les orienter vers le dispositif approprié. Ces sas ont d’ores et déjà accueilli plus de 4 000 personnes.

de l’intérieur et des outre mer. Madame la ministre, conformément à l’article 73 de la Constitution, qui prévoit la possibilité d’adapter les lois et règlements aux caractéristiques particulières des départements d’outre mer, la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a instauré un régime dérogatoire d’acquisition de la nationalité à Mayotte. Ainsi, pour un enfant né à Mayotte, il est désormais exigé que l’un de ses parents ait, au jour de la naissance, été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois. À l’heure où des voix s’élèvent pour durcir ce dispositif, il est impératif d’en connaître au préalable l’efficacité cinq années plus tard. Un bilan de la mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions d’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France des enfants nés à Mayotte de parents étrangers est il prévu ? En outre, dans son avis du 5 juin 2018 sur la proposition de loi tendant à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte les règles d’acquisition de la nationalité française par une personne née en France de parents étrangers, dont ce dispositif est issu, le Conseil d’État a souligné l’intérêt d’une campagne d’information à Mayotte et à destination des pays d’origine des personnes y immigrant irrégulièrement sur l’état du droit qui résulterait du vote de ce texte.

Elle permettrait aussi aux Français et aux étrangers en situation régulière depuis plus de trois mois de connaître les conséquences juridiques et financières encourues en cas de reconnaissance frauduleuse de paternité.

Mohamed Soilihi, comme vous l’avez souligné, la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a instauré un régime particulier pour Mayotte en matière d’acquisition de la nationalité. Cette adaptation a été prise dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, qui permet de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières

il a été décidé par le Président de la République de lutter activement contre l’immigration irrégulière en provenance de l’Union des Comores, laquelle menace de déstabiliser le fragile équilibre de ce territoire que l’un des moyens de rendre moins attractive Mayotte pour les ressortissants comoriens était de limiter l’accès à la nationalité française par le simple fait d’être né en France de parents étrangers.

l’adoption de la loi Collomb, le nombre d’acquisitions de nationalité française par des mineurs a baissé de moitié. La pression migratoire toujours plus forte nécessite de prendre des mesures plus ambitieuses, afin de ne pas laisser entrevoir la perspective d’un titre de séjour à des ressortissants étrangers du seul fait que leur enfant est né à Mayotte. Ainsi, les mesures que nous avons annoncées, au nom du Président de la République et du Gouvernement, permettront, après une révision de la Constitution, de ne plus appliquer le droit du sol à Mayotte. Le Gouvernement entend en parallèle renforcer drastiquement la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et communiquer sur ces mesures, monsieur le sénateur. En revanche, les autres modes d’accès à la nationalité, en particulier celui par décision de l’autorité publique, restent inchangés, permettant aux étrangers souhaitant acquérir la nationalité française de démontrer leur attachement à la communauté nationale et aux valeurs de la République.

premier tiers de confiance en matière de signalement de contenus en ligne illicites, l’association Point de Contact agit, depuis 1998, pour un internet sans crainte. Elle est un acteur reconnu dans la lutte contre les contenus haineux et illicites, en matière de terrorisme, de radicalisation, de harcèlement, de violences sexistes et sexuelles, de pédocriminalité. Point de Contact analyse et qualifie les informations transmises par les internautes gratuitement et anonymement, avant de transmettre ces signalements, pour retrait et

Point de Contact est l’une des neuf hotlines fondatrices de Inhope, le réseau international de lutte contre les contenus pédocriminels en ligne, qui regroupe aujourd’hui plus de cinquante pays. Les signalements opérés par ce réseau alimentent la base de données d’Interpol sur l’exploitation sexuelle des enfants dans le monde.

S’il n’existe aucun droit acquis au maintien d’une subvention, cette rupture brutale des relations établies a précipité l’association dans une impasse financière grave. Après un plan d’économies drastique, elle est à deux doigts de déposer le bilan. L’association, qui emploie quatre personnes pour éplucher des milliers de contenus illicites, réclame à l’État 41 000 euros pour éviter de mettre la clé sous la porte.

une initiative des acteurs de l’industrie d’internet, afin de permettre le signalement des contenus pédopornographiques et de haine raciale. L’association a ensuite permis à ces plateformes de répondre, pour un coût modique, aux obligations prévues par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à internet sont désormais tenus « de mettre en place un dispositif accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance les contenus illicites promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites » qui leur seraient signalées lorsqu’elles sont hébergées sur leurs serveurs et de « rendre publics les moyens consacrés à la lutte contre ces activités illicites ». Cette mission demeure l’objet principal de l’association Point de Contact. De nombreuses plateformes privées d’internet, comme Google, Facebook, Twitter, Tik Tok, ainsi qu’OVH, le premier hébergeur de serveurs français, sont aujourd’hui des adhérents de l’association.

bien été effectuée le 16 mai 2023. Compte tenu du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née à compter du 16 juillet 2023.

Selon les budgets prévisionnels de l’association, joints à sa demande de subvention pour l’exercice 2023, aucune part des cotisations versées par les acteurs de l’internet, soit 154 000 euros au total, n’est affectée à cette action. Celle ci est donc, de fait, supportée intégralement par le FIPD, à hauteur de 225 000 euros.

la journée, des jeunes filles, qui se pressent de rentrer chez elles, se font interpeller. En fin de journée et la nuit se déroulent des scènes étranges, des livraisons de colis en tout genre vers l’intérieur de la prison. Les colis sont hissés par dessus les murs de la prison au moyen de cordelettes munies de crochets, puis rattrapés depuis les fenêtres. Au début, il n’y avait qu’une seule corde ; il y en a désormais des dizaines, accrochées en permanence. Ces livraisons illicites, certains tiennent d’ailleurs à les maintenir. Leur solution : l’intimidation des riverains. J’ai en main un tract menaçant, la photo et le nom du président de l’association des riverains. Il a été placardé sur les murs de la rue Jean Dolent, et des individus se sont introduits dans les immeubles pour les glisser dans les boîtes aux lettres.

en lien avec les agents de la police municipale ; ces rondes assurent une meilleure protection que les gardes statiques. Les interventions de police sont par ailleurs facilitées par la présence de trois sites de vidéoprotection quadrillant le secteur. le secteur. Les vidéopatrouilles effectuées permettent en particulier de repérer, en amont, les comportements suspects et d’envoyer rapidement un équipage sur les lieux. Il convient de noter le lancement du projet d’installation d’une nouvelle caméra de vidéoprotection à l’angle à l’angle du boulevard Arago et de la rue de la Santé. Ces dispositifs ont permis de réduire les rassemblements de personnes aux abords du centre pénitentiaire et d’augmenter le nombre d’interpellations : 182 personnes ont été interpellées en 2023, 36 depuis le début de l’année 2024, pour des jets de colis dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire. Le commissariat du XIV arrondissement maintient un lien permanent avec les habitants et les professionnels du secteur pour une réactivité maximale des agents sur le terrain. Les policiers ont été requis à 71 reprises en 2023 et à 31 reprises depuis le début de l’année 2024. Par ailleurs, un numéro spécialement dédié aux riverains est également expérimenté depuis le 19 février dernier, leur permettant de prévenir rapidement les policiers en cas de nuisances. Il convient de souligner que ce numéro ne se substitue pas

l’est de l’arrondissement ; il regroupe notamment la direction du centre pénitentiaire et les bailleurs et syndics de copropriété, ainsi que les services de la préfecture de police, de la Ville de Paris et de la mairie d’arrondissement. voyez, madame la sénatrice, l’État est pleinement mobilisé sur cette question, au travers de ces différents dispositifs et dans un cadre partenarial, afin d’aboutir à des solutions opérationnelles pour la sécurité et la tranquillité des riverains de la prison.

concerne un secteur où la compétence en matière de circulation est partagée, la préfecture de police a émis de nombreuses réserves au regard de l’impact de ce projet sur la circulation des véhicules prioritaires, comme sur les services d’urgence, mais aussi de la complexité des modalités de contrôle qu’il faudrait mettre en place. Nous faisons face à une véritable usine à gaz qui va compliquer la vie quotidienne des Parisiens

Aussi, madame la ministre, pouvez vous nous préciser la position du Gouvernement vis à vis de ce projet qui risque de congestionner Paris ? Pouvez vous également nous préciser si la préfecture de police compte participer à la mise en œuvre et au contrôle effectif de ce dispositif ?

tandis que le préfet de police dispose, sur un certain nombre de sites, voies ou portions de voies, du pouvoir de réglementer de manière permanente les conditions de circulation. Sur d’autres axes structurants de la capitale, ainsi que sur ceux qui sont empruntés dans le cadre du déclenchement des plans de secours prévus par le décret du 18 juillet 2017, le préfet de police dispose d’un rôle prescriptif pour les aménagements de voirie projetés par la Ville de Paris. La zone à trafic limité prévue par cette dernière est un dispositif permettant de réserver certaines zones du centre de Paris aux piétons, aux vélos, aux transports en commun, aux taxis et à certaines catégories d’usagers. Le trafic de transit y sera interdit, mais le trafic de destination restera autorisé pour les usagers qui travaillent, résident ou interviennent dans le périmètre de la ZTL. Au cours de nombreux échanges, particulièrement étroits, avec la Ville de Paris, le préfet de police a indiqué à la maire de Paris que le périmètre de la ZTL ne saurait intégrer la rive gauche de la Seine, ce

d’une signalisation adaptée et une large communication sur la mesure. Tant que ces modalités ne seront pas clairement définies, le dispositif ne sera vraisemblablement ni compris ni accepté par les usagers, situation qui risque d’entraîner la congestion de certaines voies. À ce jour, le préfet de police n’a pas été destinataire du dossier complet relatif à la ZTL. Par conséquent, il ne peut pas, pour le moment, arrêter d’avis définitif sur ce sujet. En tout état de cause, la mise en œuvre du contrôle des accès

et les nuisances sonores. Madame la ministre, je veux vous dire solennellement ceci : il est encore temps que le Gouvernement s’oppose fermement à ce projet mal préparé, qui n’apportera aucune amélioration dans la capitale

qui a dû bouleverser son agenda pour retourner plus rapidement dans son département. Le 16 juin dernier, un séisme d’ampleur historique a frappé la Charente Maritime et les Deux Sèvres. Le nombre de communes reconnues en état de catastrophe naturelle s’élève désormais à Tout le monde reconnaît l’efficacité des services de l’État et de l’ensemble des services de secours au moment du séisme comme dans les jours qui ont suivi. Néanmoins, des problèmes aigus restent à régler neuf mois plus tard. Un trop grand nombre de sinistrés demeurent dans une situation de grande précarité et, surtout, d’inquiétude. Ils ont pu exprimer leur désarroi au Premier ministre lors de sa venue

Or, sans expertise adéquate, les sinistrés ne peuvent bénéficier de l’aide financière dont ils ont besoin. Des sinistrés continuent par ailleurs de rembourser leurs emprunts bancaires, alors même qu’ils doivent payer un nouveau loyer, certaines assurances ne prenant même pas en charge le relogement.

d’abord, avec le ministre de l’intérieur, à saluer les habitants des communes touchées, qui ont subi un préjudice aussi dommageable qu’imprévisible. Je remercie également, au nom du Gouvernement, les services de l’État qui se sont immédiatement mobilisés pour accompagner les collectivités et les sinistrés, sous la direction des préfets. Avec les maires, ils ont trouvé des solutions de relogement dans l’urgence, notamment la mise à disposition de mobil homes. Des centaines de familles ont bénéficié d’un suivi personnalisé et de l’appui d’une cellule consacrée au relogement.

Au delà de la reconnaissance administrative de l’état de catastrophe naturelle, les services de l’État demeurent fortement mobilisés pour accompagner les communes et leurs habitants, même après l’urgence qui a suivi

dont le but n’est pas essentiellement commercial ; elle a permis la construction d’une politique cohérente à l’endroit de ces sites, qu’ils soient protégés ou non, publics ou privés. L’ensemble de la filière était pris en compte au travers d’axes d’excellence

à leur entretien, un agrément fiscal. Il signalait à l’attention de tous et, plus particulièrement, des pouvoirs publics un lieu exceptionnel. Il apparaissait comme l’aboutissement d’un travail acharné et passionné.

acte la suppression de l’agrément fiscal, statut qui permettait en toute logique au propriétaire privé, en contrepartie d’une ouverture au public, de bénéficier de la fiscalité des monuments historiques

mais également sur les motivations qui ont poussé le Gouvernement à se désengager de toute valorisation de ces espaces, qui représentent pourtant une vraie richesse et mettent en valeur, une fois de plus, la qualité de nos territoires. Pousser les propriétaires à ne pas demander l’obtention ou le renouvellement de ce label, c’est aussi renoncer à ce que ces espaces soient largement identifiables et ouverts au grand public et priver ainsi ce dernier de l’accès à ces sites exceptionnels qui participent, comme vous le savez, au renom de notre pays.

néanmoins heureux d’apprendre que la suppression dudit agrément fiscal n’a pas découragé les propriétaires de demander ce label, puisque les demandes de labellisation sont en augmentation cette année.

Par ailleurs, en 2014, à la demande des associations de propriétaires privés, le ministère de la culture a pris contact avec la Fondation du patrimoine afin de faire bénéficier certains parcs et jardins non protégés au titre des monuments historiques des déductions fiscales offertes aux immeubles labellisés par cette fondation.

Le ministère de la culture s’est donc efforcé, tout en tenant compte de la volonté du législateur en matière fiscale comme en matière environnementale, de conserver à ce label son attractivité. territoires. Madame la ministre, la ville de Châteaurenard, située dans l’un des plus beaux départements de France, les Bouches du Rhône, est une commune historiquement agricole. Elle forme le centre d’un bassin maraîcher et arboricole de Provence depuis 1867, année de création du premier marché de producteurs de fruits et légumes. Aujourd’hui, le marché d’intérêt national (MIN) situé dans cette commune

Cela se traduira, structurellement, par la construction d’un hub composé de trois pôles. Le pôle logistique passe par la requalification de friches

ce projet d’extension du MIN de Châteaurenard, consommateur de foncier, pourra t il être considéré comme un projet d’envergure nationale afin de ne pas pénaliser la commune dans le bilan d’artificialisation des sols qu’elle devra

Les projets ne seront pas retenus en fonction de leur seul intérêt, mais tiendront compte des catégories fixées par la loi, de leur envergure significative au regard de leurs implications territoriales, ainsi que des enjeux auxquels ils permettent de répondre. Comme le prévoit la loi, le Gouvernement a porté à la connaissance des présidents de région, à la fin du mois de décembre dernier, un projet d’arrêté et une liste de projets, élaborée notamment en lien avec les préfets de région. Nous avons reçu, en toute fin de semaine dernière, l’avis du président de votre région, M. Renaud Muselier, ainsi que celui de la conférence régionale de gouvernance. Nous adresserons prochainement à M. Muselier un retour motivé sur les suites à y donner. Il pourra ensuite saisir une commission régionale de conciliation en cas de désaccord persistant sur la liste. En l’état des informations que vous me communiquez, le du projet de MIN de Châteaurenard à l’une des catégories de la loi paraît incertain, de même que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qu’il engendrerait. En tout état de cause, ce projet n’a pas fait l’objet d’une identification par le préfet de région et n’a pas été mentionné dans l’avis de la région. Néanmoins, afin de décliner la politique de sobriété foncière au plus près des besoins, présents et à venir, des territoires, le Gouvernement a souhaité que l’arrêté offre une certaine souplesse. Il pourra être révisé pour y intégrer de nouveaux projets.

une nouvelle fois, appeler l’attention du Gouvernement sur la dégradation de la ligne de train de nuit reliant Rodez à Paris, sur laquelle des incidents entraînent des annulations régulières. Depuis le 1 juillet 2023, la ligne Rodez Paris a fait l’objet de cinquante Aujourd’hui, réserver un billet sur cette ligne n’est plus l’assurance de pouvoir effectuer le trajet. Entre annulations, retards et reports de dernière minute, les usagers sont soumis à une forte incertitude.

des parlementaires de l’Aveyron et le maire de Rodez, afin d’envisager des solutions et des perspectives. C’est pourquoi j’attends, avec tous les Aveyronnais, des réponses précises. Madame la ministre, le Gouvernement va t il développer le parc de matériel roulant et investir dans de nouvelles locomotives ? Va t il doter les centres de maintenance de plus de moyens ?

Les annulations qui ont eu lieu à la fin de l’année 2023 sont essentiellement dues à des difficultés de maintenance des locomotives diesel qui tractent les voitures entre Brive la Gaillarde et Rodez. En effet, ces derniers mois, de nombreux incidents sur les voies ont entraîné une surcharge dans les centres de maintenance habituels. L’État, en tant qu’autorité organisatrice des trains de nuit, a financé la location d’une locomotive supplémentaire à Brive la Gaillarde, qui vient renforcer le parc de locomotives utilisé pour les dessertes de Rodez, Albi et Aurillac. Les recherches de locomotives supplémentaires se poursuivent en parallèle. Forts du constat Forts du constat que le matériel actuellement utilisé est ancien et ne répond plus aux attentes des usagers en matière de service, de confort et d’accessibilité, les services de l’État travaillent sur des modalités de renouvellement. Par ailleurs, l’État investit massivement dans l’infrastructure ferroviaire. En particulier, la ligne Paris Orléans Limoges Toulouse bénéficie, en complément de son programme de régénération, d’un programme de modernisation dans lequel l’État investit 257 millions d’euros.

les incinérateurs ne sont pas inclus dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, seules des obligations de récupération sont prévues. De manière plus générale, les émissions de gaz à effet de serre de la gestion des déchets représentent près de 3 % des émissions nationales, soit environ 13,5 millions de tonnes de CO2 en 2023. Une grande partie de ces émissions sont liées à la mise en décharge, le méthane et le protoxyde d’azote ayant des pouvoirs de réchauffement global plus importants que le dioxyde de carbone. La récente révision du marché carbone européen a introduit de nouvelles obligations. Pour les incinérateurs, elles se limitent, à partir de 2024, à une surveillance et à une déclaration des émissions de gaz à effet de serre des installations. À ce stade, la réglementation européenne ne prévoit pas d’obligation de restitution de quotas carbone, donc l’application d’un prix carbone pour les incinérateurs. Les déchets sont néanmoins utilisables dans l’industrie, soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, notamment sous forme de combustible solide de récupération. la directive prévoit une clause de revue d’ici au 31 juillet 2026. À cette échéance, la possibilité d’inclure pleinement les incinérateurs dans le système d’échange de quotas

de la Commission européenne, ainsi qu’une discussion entre colégislateurs. Si cette proposition aboutit, le Gouvernement sera attentif aux implications économiques pour les incinérateurs et les collectivités. terminé avec les réponses à des questions orales. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de de la filière nucléaire et du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010 837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ont été publiées.